que si les exploitations sont économiquement viables. Nous avons bien conscience que, par définition, la recherche de la viabilité économique est une condition majeure, voire indispensable, pour qu’un projet d’installation soit mené à bien. Cette réalité s’impose d’ailleurs dans quasiment tous les pans de notre économie. Toutefois, nous avons également conscience que les rapporteurs de notre commission des affaires économiques ne sont pas très enthousiastes quand il est question de transition agroécologique ou de soutien à l’agriculture biologique.

pour l’alinéa 28 : il s’agit de « favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique au sens de l’article L. 13 du code rural et de la pêche maritime, et un développement de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique en adéquation avec la demande de ces produits, en réduisant les importations de ces produits et et en développant l’appareil industriel de transformation agroalimentaire pour diversifier l’offre et répondre au mieux à la demande ». Voilà

bio fournit la preuve que c’est complètement l’inverse. Si votre production n’a aucune compétitivité, vous n’avez aucune souveraineté.

Cela ne vaut pas que pour les produits agricoles : ce système est global. Dire que compétitivité et souveraineté sont antinomiques, c’est mettre à mal les bases mêmes

mettre la pression ! Monsieur le sénateur, vous n’ignorez pas le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales

près de la moitié des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite d’ici à 2030. Si nous n’agissons pas, c’est tout notre modèle agricole, nos territoires ruraux et notre souveraineté alimentaire qui seront fragilisés. Les espaces tests agricoles une réponse concrète à ce défi. Ils permettent aux futurs agriculteurs, y compris à ceux qui ne sont pas issus du monde agricole, de tester leur projet en conditions réelles, de se former et de tisser des liens avec les cédants. d’un outil précieux pour assurer la transition des exploitations et encourager une agriculture durable, locale et diversifiée. Un tel dispositif a donc toute sa place dans une loi censée favoriser le renouvellement des générations en agriculture. Il convient donc de le

Cet amendement vise à souligner l’importance du maintien de l’élevage durable français. Pour assurer le maintien de cet élevage de qualité, qui fait l’exceptionnalité du modèle agricole français, il est nécessaire d’assurer l’approvisionnement en produits issus de ces élevages de tous les lieux de consommation, notamment

En conséquence, les filières bovine, porcine et avicole françaises durables, notamment celles en agriculture biologique et en plein air, peinent à se maintenir. La part des poulets standards progresse : elle représentait 72 % de la production en 2023, contre 65 % en 2020. l’enjeu n’est pas tant un déficit en volume de viande qu’une stagnation de l’offre durable et des débouchés associés, faute d’une réelle politique alimentaire et en raison d’un développement non régulé de la consommation hors domicile.

Nous sommes bien évidemment favorables à cette disposition qui participerait pleinement et de manière même plus ambitieuse à l’objectif fixé dans le plan Protéines végétales, consistant à doubler la part de SAU consacrée à ces cultures, pour atteindre 8 % en 2030. Les légumineuses sont un enjeu stratégique pour notre agriculture si nous souhaitons répondre aux défis que nous aurons à affronter dans les décennies à venir. Les crises de ces dernières années, qu’elles soient sanitaires ou diplomatiques, ont démontré la fragilité de notre modèle, trop dépendant des importations. Nous devons donc retrouver au plus vite notre autonomie et notre indépendance dans de nombreuses filières, dont celle des légumineuses. C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d’adopter une attitude volontariste face à ces

doit rester un simple complément à l’activité agricole et qu’elle ne saurait se substituer à la vocation fondamentale de l’agriculture, qui est de produire de la nourriture.

Nous abordons ici un sujet sensible et souvent clivant. Pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, la vocation première de l’agriculture est de nourrir la population et elle doit absolument le rester. Nous pouvons entendre que, dans certaines situations, la production d’énergie, si elle reste secondaire, peut constituer une source de revenus complémentaires bienvenue pour les agriculteurs. Mais si, dans ce cadre restreint, qui doit être fermement réglementé, notre agriculture peut participer à la production énergétique, elle ne peut pas en faire une priorité. De plus, nous savons tous que la question de la production d’énergie sur les exploitations agricoles est source de spéculation foncière, qui affectera nécessairement les générations futures. Les jeunes se trouvent déjà parfois dans l’incapacité financière d’acquérir du foncier… Le présent amendement vise donc à inscrire noir sur blanc dans la loi que le concours apporté par l’agriculture à la transition énergétique de la Nation ne peut en aucun cas remettre en cause sa vocation première, qui est la production alimentaire.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à orienter les politiques publiques de recherche, d’innovation et de développement vers les pratiques agroécologiques.

robotique, numérique, génétique », de favoriser l’endettement et de privilégier les plus grandes exploitations, nous sommes convaincus que les pratiques agroécologiques, moins coûteuses et validées par la science, sont bien plus bénéfiques pour les agriculteurs

Les agriculteurs eux mêmes ne cessent de le répéter. Le sol est un agent essentiel de la régulation du climat, au travers de ses multiples services écosystémiques, du cycle de l’eau à la fertilité des océans, de notre alimentation à la captation du carbone. une étude de 2023, 98 % des terres agricoles françaises sont contaminées par au moins une substance phytosanitaire. Cette dégradation des sols réduit leur capacité de séquestration du carbone.

enjeux relatifs à la brevetabilité du vivant et à l’accaparement de ce dernier par de grandes multinationales semencières. Nous avons pu constater que notre amendement a suscité une levée de boucliers de la part d’une partie bien précise du monde agricole, qui s’est fendue d’un courrier pour en dénoncer la portée.

en agriculture, incluant la protection contre l’ensemble des aléas climatiques, sanitaires et environnementaux. Ce dispositif garantirait une couverture équitable pour tous les agriculteurs, renforçant par là même la résilience et la solidarité nationale.

a été déployée, dotée d’un budget important et inédit de 680 millions d’euros par an. Ce nouveau dispositif est plus attractif et permet, quand il fonctionne convenablement, à chaque exploitant d’accéder à une couverture assurantielle renforcée.

Les impacts négatifs de la spécialisation des territoires sont nombreux : pollutions de l’eau, algues vertes dans les régions excédentaires en élevage – je connais particulièrement ce sujet –, difficultés à développer des systèmes alimentaires territorialisés, ou encore recours accru à des intrants de synthèse. Favoriser une diversification des activités agricoles dans les territoires, en particulier une meilleure répartition spatiale des activités d’élevage, ainsi qu’une complémentarité renforcée entre productions animales et végétales, est une nécessité pour améliorer la souveraineté alimentaire et assurer la transition écologique de l’agriculture. La redistribution spatiale des activités d’élevage doit être planifiée et accompagnée. Cela permettrait de poser la question des besoins infrastructurels et techniques indispensables à sa réalisation au niveau des territoires, à la fois en termes qualitatifs – compétences, fonctions – et quantitatifs – nombre d’emplois ou d’infrastructures nécessaires. Une planification par des acteurs publics, mais aussi privés, est déterminante pour définir une trajectoire et assurer les moyens nécessaires : je pense à des expérimentations de restructurations diversifications de fermes, ou encore au financement d’outils de transformation, notamment d’abattoirs locaux. Lors des concertations mises Lors des concertations mises en place en vue de l’élaboration de ce projet de loi, la question de la diversification avait fait l’objet d’un consensus. Les politiques publiques doivent donc accompagner cette déspécialisation tout en veillant à prendre en compte les spécificités. Quel est l’avis de la commission ? Il est défavorable,

tantôt des terres de grandes cultures dans l’Hexagone, tantôt un modèle familial sur nos territoires ultramarins. D’ailleurs, dans nos outre mer, nous observons uniquement des exploitations de petite dimension, avec une surface moyenne de 5 hectares, contre 69 hectares pour la moyenne des exploitations hexagonales. Ces exploitations sont, chez nous, évidemment structurées autour d’un équilibre parfois fragile entre les filières de diversification et les filières historiques d’exportation, à savoir la canne à Il nous faut aujourd’hui admettre la singularité des réalités locales, notamment dans les politiques publiques. Ne pas prendre en compte les évidentes particularités géographiques et climatiques des territoires ultramarins, c’est empêcher le développement de modèles économiques agricoles. Alors même qu’il s’agit ici d’un programme non pas hexagonal, mais bien national, il est indispensable de mentionner spécifiquement dans le texte, à l’alinéa 33, aux côtés des zones de montagne et des zones dites « intermédiaires », nos départements et régions d’outre mer. Je vous invite donc, au travers de cet amendement, à consacrer les singularités et la diversité de l’ensemble de notre beau territoire national. Quel est l’avis de la commission ? Cet

il est bien précisé : « La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre mer ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. comme finalité aux politiques publiques « d’assurer, à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État

proposons que soit spécifiquement encouragé le développement des labels agricoles, qui sont l’une des clés de la recherche de la souveraineté alimentaire. Ces labels participent à la diversification et à la valorisation de nos productions et de nos territoires. À ce titre, ils sont indispensables à une production agricole harmonieuse et de qualité.

n’y fait pas non plus expressément référence, évoquant plutôt toutes les productions sous signes de qualité et d’origine. Nous proposons donc de remédier à cet oubli regrettable et de reconnaître spécifiquement les labels de production agricole au sein de l’article L. 1

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à renforcer la définition de la souveraineté alimentaire en insistant sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail, les revenus et la protection sociale des agriculteurs, ainsi qu’en luttant

Il convient également d’améliorer la protection sociale, dans un contexte où les retraites agricoles sont extrêmement faibles, en particulier pour les femmes, et où les agriculteurs rencontrent des difficultés à accéder au remplacement en cas d’arrêt maladie ou de congé de maternité ou de paternité. Il convient notamment d’agir, à ce titre, sur la prise en charge des maladies professionnelles. il faut améliorer les conditions de travail des agriculteurs, notamment face aux risques d’épuisement professionnel et d’isolement. En particulier, il convient de lutter contre les risques

le risque de mortalité par suicide restait en 2020 supérieur de 77,3 % à celui des assurés tous régimes confondus. Tous ces éléments doivent donc nous amener à apporter une attention particulière à la santé des agriculteurs.

le Gouvernement depuis des années sur le manque d’efficacité des lois Égalim, qui ne vont pas assez loin dans la coercition pour imposer à certains acteurs économiques de changer leurs pratiques, destructrices pour les agriculteurs.

que les marges de l’agrobusiness, qui tient la FNSEA, soient préservées. Il le sait et l’explique parfaitement, et pourtant, d’amendement en amendement, il nous propose d’aller toujours plus loin dans l’impasse. Bravo !

Il y a quelques dizaines d’années, un médecin de campagne s’installait seul dans son cabinet ;

madame la ministre,

une jeunesse qui ne demande qu’à s’engager dans ce magnifique métier du vivant.

négociations commerciales » au profit des producteurs pour assurer un meilleur équilibre des relations commerciales. Cet ajout est fondamental pour permettre aux producteurs de défendre leurs intérêts face à l’aval et de leur assurer une plus juste rémunération au moment des négociations commerciales.

est à Mme la ministre. C’est un amendement auquel j’attache une importance toute particulière. Il a pour objet la valorisation du rôle des agricultrices

comme illustration les effets de la fluctuation des marchés mondiaux sur la compétitivité des filières sucre et banane, ou encore des événements majeurs tels que les ouragans ou les cyclones, comme celui qui a frappé à Mayotte tout récemment.

Cette moyenne ne reflète cependant pas la diversité des situations dans nos territoires. À La Réunion, le taux de couverture des besoins de la population par la production locale dépasse ainsi 70 %.

nous estimons qu’il doit d’abord permettre d’orienter les filières et d’accompagner les agriculteurs, notamment ceux qui souhaitent tendre vers des modèles durables et résilients d’un point de vue socioéconomique et environnemental. amendement tend à réorienter les objectifs du plan stratégique pour les rendre plus ambitieux d’un point de vue agroécologique. Nous proposons également d’assurer le maintien de l’élevage dans les systèmes de plein air, herbagers et biologiques, et d’accompagner la transition de l’élevage français vers ces systèmes,

de mon point de vue, indispensables à la bonne santé de l’organisme. Aussi convient il de maintenir l’ensemble des fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales de l’élevage, ainsi que ses complémentarités agronomiques

pour lesquels nous disposons de données et qui rendent compte des besoins alimentaires en France. Les taux de couverture de la consommation par la production nationale et la dépendance aux importations sont déjà calculés et publiés par FranceAgriMer – j’en ai parlé

veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole, notamment en allégeant la fiscalité sur l’énergie, dont le carburant, » – je vous renvoie

compte du principe d’annualité budgétaire et de la nécessité d’adapter nos outils fiscaux à la réalité économique de l’agriculture.

Une mission visant à étudier les options possibles pour indemniser les producteurs en agriculture biologique touchés par des destructions de lots et des déclassements va être confiée conjointement à l’inspection générale des finances l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd) et au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.

et ils conservent nos paysages et notre souveraineté alimentaire. Les élevages moins autonomes sont plus dépendants des intrants et peut être plus fragiles.

qui sont tout à fait favorables à l’alimentation.

même si la Commission européenne doit les valider. Nous pensons tout particulièrement au Pacte vert européen et à la stratégie « de la ferme à la table ». Au cours des dernières années, les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont dénoncé à plusieurs reprises le manque de transparence et de dialogue

Notre amendement vise donc à accélérer la mise en œuvre effective des objectifs stratégiques de développement de l’agriculture ultramarine, en ciblant l’impératif de souveraineté alimentaire. Les agriculteurs d’outre mer

cette fin, nous souhaitons que, chaque année, le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant « les perspectives de développement de chaque filière et faisant état de l’évolution du revenu agricole, de la part de foncier arable disponible, du nombre de transmissions et renouvellements d’exploitations réalisés dans l’année, du nombre de formations dispensées, de l’état écologique des milieux et des pratiques agraires à encourager pour maintenir une haute exigence environnementale